La séance est ouverte. Le comprendre analytiques de la précédente séance a été distribué, il n'y a pas d'observation, je n'en vois pas donc le procès verbal est adoptée sous les réserves d'usage. En application du 5ème alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique et de la loi du 13 juillet 2010 prises pour son application, la commission des finances, a émis un avis favorable 20 voix pour, une voix contre et 4 bulletins blancs à la nomination de Monsieur Éric Lombard aux fonctions de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. la parole est à monsieur Loïc Hervé pour une mise au point sur un vote. pour la séance du 28 novembre 2017 portant sur l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances, formule 18 et lors de ce scrutin Madame Sophie Joissains souhaitaient s'abstenir je vous remercie. Très bien acter donner de votre mise au point pour le compte de madame Sophie Joissains cette mise au point, sera publié au Journal officiel et figurera dans l'analyse politique du scrutin. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances adoptées par l'Assemblée nationale pour 2018. Nous commençons l'examen au sein de la seconde partie du projet de loi de finances des différentes missions. Le Sénat va examiner les crédits de la mission, relations avec les collectivités territoriales et article 58 62 bis et du compte spécial avance aux collectivités territoriales, donc la parole est à monsieur Charles Denner, rapporteur spécial de la commission des finances. Monsieur Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Bien que nous examinions ce ce matin, les crédits de la mission, relations avec les collectivités territoriales et et du comte de concours financier avance aux collectivités territoriales, il me semble indispensable de replacer cette mission dans le contexte plus global des finances locales, en ce qui concerne la loi de programmation des finances publiques, le Sénat a considéré que la trajectoire de réduction de dépenses proposées par le gouvernement revenait à demander aux collectivités territoriales de réaliser 21 milliards d'euros d'économies, et non 13 milliards d'euros, comme il l'indique. La relation de confiance entre l'État et des collectivités territoriales, prônée par le gouvernement, a ainsi été écornée d'entraide je dirais-je en première partie du présent projet de loi de finances, le gouvernement a proposé de supprimer sur 3 ans, la taxe d'habitation pour 80 pourcent des Français, le Sénat a considéré que cette réforme qui ne répond qu'imparfaitement à la question des inégalités liées à l'obsolescence des valeurs locatives n'étaient pas mûrs et qu'il convenait de la reporter en effet les valeurs locatives obsolète et injuste continueront à être utilisées pour établir la taxe d'habitation de 20 pourcent des contribuables, mais aussi la taxe foncière ou ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères outres les injustices entre contribuables qui soulève d'ailleurs un risque contentieux : l'absence de révisions entraîne des injustices entre collectivités territoriales puisque les valeurs locatives sont utilisés dans les dispositifs de péréquation, par le biais du potentiel fiscal qui mesure leur richesse relative il nous appartiendra collectivement de définir un nouveau cadre des finances locales en s'attaquant à la fois à la réforme de la fiscalité des dotations et de la péréquation dans cette perspective, nous envisageons de vous proposer lors de l'examen des articles non rattachés un amendement visant à élargir à l'ensemble des départements l'expérimentation sur la révision des valeurs des bases locatives menée par la DG Philippe dont les conclusions ont été présentées au parlement au début de l'année 2017 ce préalable indispensable à la révision permettrait au législateur de décider, le cas échéant des dispositifs à mettre en oeuvre pour atténuer les transferts de charges entre contribuables. Sur un plan plus général, nous pensons qu'au-delà des dispositions purement technique de ce PLF qui ont un côté un peu frustrant, nous sommes à la croisée des chemins et il convient que, effectivement, ainsi que le propose le président de la République de préparer une réforme globale de la fiscalité locale à l'horizon 2020 après la suppression de la TP hier TH demain le système imaginé il y a un demi-siècle et sur les mécanismes duquel nous vivons perd c'est 2 6, ses 2 pieds et doit être totalement reconsidérés pour ce faire, il faut avant toute chose, repenser les fondamentaux des finances locales et publiques à l'aune des modifications profondes intervenue dans notre pays et au plan mondial, lesquels en ont radicalement modifié l'écosystème la territorialisation de l'impôt n'est plus compatible avec la christianisation géographique de l'économie et l'urbanisation de la population, l'appréhension des charges au niveau communal à l'aide d'indice synthétique assis sur l'habitant ne répond plus aux défis du retrait des services et des acteurs publics, de la ruralité, une nouvelle prise en compte de la centralité s'impose, celle des standards italiens que nous avons étudier avec Claude rénal nous apparaît innovante et intéressante une nouvelle gouvernance systémique des finances publiques doit être également être mis en place permettant à la fois nos métropoles d'assurer leur compétitivité internationale et aux territoires d'être servi équitablement afin de réduire la fracture qui s'est ouverte et, le cas échéant de contribuer au financement de la dette nationale, il est urgent de faire partager au plus vite des fondamentaux d'une telle réforme avant d'en décliner les mécanismes en toute lisibilité dans une approche probablement de la décentralisation et de la libre administration des collectivités plus contemporaine, les sénateurs, dont 7 corps de métiers sont prêts à apporter leur part dans cette réflexion, puis leur technicité dans la vie 09 de ce défi, une coproduction de la réforme participerait de la confiance réclamé et des prémices de cette nécessaire gouvernance partagée, voilà pour le cadre global en ce qui concerne les crédits de la mission, relations avec les collectivités territoriales en 2018 les autorisations d'engagements prévus sur la mission diminue de 12 pourcent soit 524 millions d'euros, essentiellement en raison de la non-reconduction du fonds exceptionnel destiné aux régions et de la suppression de la réserve parlementaire, madame la ministre, lors de votre présentation du projet de loi de finances pour 2018 devant notre commission des finances, vous avez indiqué que les subventions d'investissement aux collectivités territoriales atteindront en 2018, 1,8 milliards d'euros, soit une augmentation de 5,5 pourcent à structure constante, nous contestons cette présentation qui consiste à comparer la nouvelle dotation de soutien de l'investissement local décide qui comprend les contrats de ruralité et l'enveloppe venus se substituer à la réserve parlementaire avec l'ancienne décide qui ne comprenaient ni la réserve parlementaire ni les contrats de ruralité nous notons au contraire une diminution de ses subventions d'investissement de de son 11 millions d'euros, soit une réduction de plus de 10 pourcent par rapport à la dernière afin de soutenir les collectivités territoriales, le Sénat a adopté lundi lors de l'examen de la première partie du projet du projet de loi de finances, l'amendement que j'ai cosigné avec Claude rénal rétablissant les crédits manquants de la réserve, la réserve parlementaire destinée aux collectivités territoriales, soit 36 millions d'euros grâce à la création d'un prélèvement sur recettes spécifiques. Hormis les subventions d'investissement de Tr des PV cils, la plupart des crédits de la mission, relations avec les collectivités territoriales correspondent à des compensations de transferts de compétences, la commission des finances, a donc décidé de donner un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission, relations avec les collectivités territoriales, par ailleurs, c'est par le compte de de concours financier avance aux collectivités territoriales que transitent les impositions locales versée mensuellement par l'État en collectivités territoriales 107,1 milliards d'euros sont prévus à ce titre pour 2018, la commission des finances, a donc décidé de donner un avis favorable à l'adoption des crédits de ce conte de concours financiers, je vous remercie pour votre attention. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais revenir d'un mot sur les propos de mon collègue à l'instant, Charles et sur le dégrèvement 2018 d'un tiers de la taxe d'habitation, si la commission des finances, a effectivement souhaité reporter d'un an, cette réforme, je considère pour ma part, que les conditions de sa mise en oeuvre en 2018, permettre d'y être favorable, se réserve qu'elle soit entièrement neutre pour les collectivités locales et que 2018, cela a été dit, soit mise à profit pour rechercher les termes d'une remise à plat du financement des collectivités locales, tant du point de vue fiscal que des dotations ou des nécessaire péréquation par ailleurs je souhaiterais compléter le cadre général présenté par mon collègue Charles Denner en soulignant que si, comme le répète le gouvernement, la dotation globale de fonctionnement ne diminue pas en 2018 c'est un drôle de pacte qui est toutefois proposée aux collectivités territoriales la première lecture au Sénat du projet de loi de programmation des finances publiques a permis de clarifier et de corriger le texte, néanmoins, de nombreuses zones d'ombre demeurent, nous ne savons toujours pas quel sera finalement la marge de manoeuvre réelle de négociations auront les préfets dans leurs discussions avec les collectivités territoriales ou si l'effort sera fait en fait réparties selon des critères précis, nous ne savons pas non plus quels critères seraient alors évidemment utiliser nous avons lu quelques propositions assez général finalement de la mission d'Alain Richard et Dominique Bur sur le sujet assez générale à ce stade, se pose également la question du périmètre des collectivités qui hériterait alors concernés par la contractualisation les plus peuplées, comme le propose le projet de loi de programmation ou les plus importantes, financièrement, comme semble le suggérer la mission Richard Burr, par ailleurs, nous ne savons pas quand les collectivités connaîtront l'objectif qu'il aura sera signé pour 2018, le temps que les différents organes de réflexion et de concertation est achevé leurs travaux le risque et qu'on leur assigne à l'été seulement des objectifs sur leurs dépenses 2018 sur le respect des quelles pourraient être sanctionnés éventuellement quelques mois plus tard, enfin la pente de croissance des dépenses pour l'instant retenu de 1,2 pourcent en valeur et en moyenne, soit quelque chose de lors de l'inflation, au mieux, n'augure rien de bon pour les collectivités qui seront soumises, je vous rappelle que nous avions étudié en 2015 avec Charles Guené, les modalités d'associations, des collectivités territoriales à la maîtrise des finances publiques en Autriche et en Italie, ce travail pourrait aujourd'hui se révéler fort utiles en particulier la pertinence et l'objectivité des critères de ressources et de charges utilisées pour répartir les concours financiers de l'État et la péréquation sont fondamentales, si l'on souhaite que cette répartition soit véritablement juste nous vous proposerons tout à l'heure, un amendement visant à étudier la mise en place d'un système inspiré des besoins de financement standard italien je voudrais également abordé le sujet de la minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle dessert prévue par le projet de loi de finances, elle le symptôme d'un système à bout de souffle, le gouvernement se réjouit que les minoration historiques voient désormais leur taux de compensation, joli, il se trouve que Madame la Ministre, vous n'aviez plus le choix parce qu'il ne reste quasiment plus rien, elles représentent au total 57 millions d'euros après avoir été minoré de près de 800 millions de Roland Garnier et 200 à 300 millions d'euros chacune des années précédentes, vous avez donc été contraint de vous rabattre sur la desserte épée une dotation destinée à compenser à l'Euro près les perdants de la réforme de la taxe professionnelle de 2010, auxquelles on avait bien entendu jurer qu'il s'agissait d'une compensation pérenne ce faisant vous attaquez à des territoires qui sont souvent déjà en perte de vitesse à d'anciens territoires industriels et vous préserver totalement des collectivités parmi les plus riches, mais en même temps je corrige, puisqu'on a vu arriver ce matin en commission un amendement du gouvernement qui, peut-être, pour M. Haute modifier cette vision sur ce sujet également, je vous invite à vous plonger dans le rapport de 2016 que nous avions commis également toujours avec mon collègue Charles Denner sur la réforme de la DGF nous proposions un système qui a pu sans doute apparaîtront peu complexe qui permettait de repartir sur des bases beaucoup plus saine, nous proposions dans ce même rapport, de modifier le fonctionnement de l'écrêtement de la dotation forfaitaire, nous pouvons nous réjouir que les dispositions adoptées l'an dernier, qui reprenait cette idée et permis d'être à passé la part des communes écrêter de 60 pourcent à 13 pourcent alors même que le montant de l'écrêtement augmenter de plus de 40 ainsi la participation au financement de la hausse de la péréquation est reparti d'une façon beaucoup plus juste, en tout état de cause, cette réforme est encore devant nous je souhaiterais que le ministre nous dise comment le gouvernement envisage de lancer les travaux concrets de la réforme de la fiscalité locale, bien sûr, suite aux travaux de la mission Richard en l'attente un moratoire sur l'ensemble des éléments constitutifs notamment des éléments de péréquation serait semble-t-il mais chers collègues souhaitables, enfin, s'agissant des crédits de la mission et du conte le concours financier j'invite à mon tour le Sénat les adopter les rejeter d'ailleurs conduirait tout simplement à priver les collectivités territoriales de 3,8 milliards d'euros de dotations versées par l'État, ce que je ne vous suggère pas, je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur, la parole est à monsieur Loïc Hervé, rapporteur pour avis de la commission des lois.

la commission des lois, comprend les raisons qui conduisent nos collègues des Finances a demandé l'adoption des crédits de la mission, relations avec les collectivités territoriales, ce n'est évidemment pas pour couper les vivres aux collectivités, mais pour exprimer vigoureusement sa préoccupation sur l'évolution de leurs ressources et de l'aide du principe de l'autonomie financière à la lumière de ce projet de loi de finance d'ailleurs comme du projet de loi programmation des finances publiques exprimé notre préoccupation, c'est d'ailleurs à peu près tout ce que nous pouvons faire, étant donné les règles de la discussion budgétaire qui corps le pouvoir d'initiative du Parlement la mission RCT elle-même est marquée par des évolutions contrastées, les dotations de décentralisation destinées à compenser les charges transférées aux collectivités sont gelés depuis 2009 et leur allant érosion due à l'inflation se poursuivra l'an prochain en 10 ans, elles ont perdu près de 9 pourcent de leur valeur réelle s'agissant des dotations d'investissement, le gouvernement assume les engagements passés mais il réduit la voilure pour les années à venir, puisque les autorisations d'engagement diminue elle de près de 13 si l'on peut saluer la pérennisation de la dotation de soutien à l'investissement local South affichée masque d'importants changements de périmètre on outre et dotation d'investissement librement distribuées par les préfets viennent peu à peu se substituer aux ressources dans les collectivités disposent en propre pour investir les nouvelles règles prévues par le projet de loi de programmation ne feront graver cette tendance contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales, les élus locaux, au travers de leurs associations représentatives nous l'ont dit, la il est un outil de recentralisation, c'est pourquoi la commission des lois a déposé plusieurs amendements pour renforcer le rôle à la fois des parlementaires et des élus locaux dans l'attribution des subventions d'une manière plus générale, la commission des lois, s'inquiète pour l'autonomie financière des collectivités territoriales, qui est l'un des piliers de notre droit de la décentralisation, la réforme de la taxe d'habitation fait planer de lourdes incertitudes sur les communes et les intercommunalités si le mécanisme du dégrèvement préservent leurs ressources et leur pouvoir de taux, le gouvernement envisage expressément de supprimer ou de limiter ce pouvoir de taux à l'avenir, j'espère d'ailleurs, Madame la Ministre, que vous pouvez nous répondre et apporter des éclaircissements sur ce sujet précis, plus largement, l'autonomie financière des collectivités territoriales est mise à mal par la disparition progressive des impôts locaux et leur remplacement par des impôts nationaux transféré sur lesquels nos collectivités n'exerce en général plus aucun pouvoir de taux ou d'actions, la différence entre la fiscalité transférée et dotation est largement surestimé, ce qui n'est d'ailleurs n'est pas le cas dans d'autres pays européens, tout cela tient au fait que la notion de ressources propres des collectivités a été défini de manière très large, trop large, peut-être par la loi organique de 2004, il faudra un jour réfléchir à sa modification, c'est donc sous le bénéfice de ces observations que votre commission des lois a donné un avis défavorable à l'adoption des crédits de cette mission. Merci dans la suite de notre discussion, je vous rappelle que le temps de parole attribués à chaque groupe pour chaque unité de discussion qu'on prend le temps d'intervention en général et celui de l'explication de vote par ailleurs le gouvernement dispose au total de 20 minutes pour intervenir. Donc la parole et, dans cette discussion est à monsieur Alain Marc, pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la ministre. Messieurs les rapporteurs. Mais, chers collègues, ce projet de loi de budget joint au projet de loi de programmation des finances publiques pour les emmener 2018 à 2022. Témoignent d'une grande défiance vis-à-vis des élus locaux, alors même qu'il faudrait à l'évidence : essayer de rétablir la confiance. Les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales subissait, c'est une nouvelle baisse. En volume, qui atteindra 5 pourcent au terme de la programmation quinquennale. Les dotations d'investissement relevant de la mission en relation avec les collectivités territoriales connaît 30 Delaney prochaine une diminution conséquente à l'autorisation de management masqué dans le projet de loi par des effets de périmètre cette baisse atteint 29 pourcent même volume pour la seule notation de soutien à l'investissement local. Oui, l'État est dans une situation de défiance à l'égard des collectivités, il y a aussi des comportement insidieux comme la ponction de près de 200 millions d'euros sur les agences de l'eau ces dernières accompagner les communes qui, conformément à la loi sur l'eau souhaitera rendre au milieu naturel une eau assainie, or les programmes d'aide aux communes risquent de ce fait d'être retardés ou d'être moins conséquent diminuant d'autant la capacité d'auto-financement des communes. Le projet de loi de programmation des finances publiques pour la période 2018, 2022 prévoit un effort de réduction des dépenses publiques des collectivités de 13 milliards d'euros en 5 ans efforts extrêmement importants alors qu'elles ont déjà réalisées, les économies qui leur était fixé lors du mandat précédent. Je précise que les collectivités locales sont les seuls à respecter les contraintes budgétaires dès lors pourquoi les étouffer leurs dettes ne représente que 10 pourcent dès 2002 ça milliards d'euros de dettes nationales et nous savons qu'elle sera forcément remboursés, puisque les Budgets sont votés à l'équilibre, on entretient l'idée que les maires seraient de mauvais gestionnaire, on les prive de leur autonomie et même anglais infantilise pour ma part, je fais confiance aux élus locaux qui ont tracé des trajectoires vertueuse en réduisant leurs dépenses de fonctionnement pour se ménager des possibilités d'investissement, que se passera-t-il pour je j'à l'Aveyron, par exemple le conseil départemental a réduit notoirement son personnel pour continuer d'investir et nous investissons à peu près 40 millions d'euros par an sur les routes, ce n'est pas rien, d'autant que dans le BTP, 62 pourcent de investissements et de l'investissement public. Et le président requis me dit qu'on a de belles routes, je suis très heureuse cette émission budgétaire précisément ignore ostensiblement le département, or les départements rassure pour le compte de l'État sur leurs propres deniers 3 allocations individuelles de solidarité la PCH a pas et le RSA tout en me faisant face à la division par 2 du fonds d'urgence doté de 200 millions d'euros. Chacun s'accorde à reconnaître que la situation financière d'une grande majorité de de pas de départements, les critiques toutefois aussi solution n'est esquissée et nous nous dirigeons vers l'accentuation de la fracture territoriale entre la France et périphérique et celle des métropoles pour revenir à l'échelon communal, l'attribution de la des TRA dépendent du bon vouloir des préfets, c'est la raison pour laquelle je souhaite nous sommes nombreux ici à souhaiter que l'ensemble des députés et sénateurs participent aux commissions départementales et que la vie de celle-ci s'pas au préfet. Concernant le seuil à partir duquel la commission de la NAVY sur les projets proposés, il serait pertinent de l'abaisser, avait 1000 euros 50000 euros, c'est beaucoup trop SAMU aussi on sait très bien que dans nos petites communes et nos communes rurales ou de villes moyennes, hé bien, nous avons des projets qui sont souvent aidés pour 40000 50000 euros, donc à des sols, ce seuil avait 1000 euros j'ai ainsi déposer des amendements en ce sens, il est un effet particulièrement l'important de renforcer le rôle des élus nationaux sur le territoire, d'autant plus que la disparition de la réserve parlementaire les a privés de moyens de soutenir des proches, des petits projets locaux qui n'aurait pas bénéficié par ailleurs de subventions état juste un exemple, je me rappelle, lors de la com bagne électorale des sénatoriales de 2014, nous sommes passés dans une commune

également nécessaire d'abaisser le seuil d'éligibilité de TER de la det qui donnera, je cours pour les petites communes, pour conclure, je voudrais profiter de s'être Tribune pour rendre nos hommage appuyé à tous les maires des petites communes rurales et les autres, ces élus exemplaire qui ne comptent pas leur temps pour rendre service à leurs administrés qui s'engage au quotidien pour dynamiser leur territoire pour créer du lien avec bien souvent hélas peu de moyens, je veux ici saluer leur engagement au service de l'intérêt général, madame la ministre mais, chers collègues, les élus locaux, les maires n'ont que faire des déclarations d'amour à leur égard, ce qu'ils veulent désormais ce qui valent ce projet de loi de budget ne répond ni aux besoins ni aux attentes de nos collectivités territoriales, bien au contraire, il dessine des perspectives très préoccupante, non seulement pour leurs ressources et leur autonomie financière, mais également pour l'investissement local aussi le groupe les indépendants ne votera pas les crédits de la mission en relation avec les collectivités territoriales du projet de loi de finances pour 2018. Donc, la parole est à monsieur Éric Gold pour 6 minutes. Monsieur Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, Lorsque l'on aborde l'examen de la mission, relations avec les collectivités, on sait pertinemment que l'on a, ce faisant, qu'une vision partielle de ces rapports, qui ne sont pas du point de vue des élus, marquée par une confiance régulière et aveugle, les 3,78 milliards d'euros inscrit en autorisations d'engagement dans cette mission, en diminution de 12 pourcent doivent être mises en regard avec les plus de 48 milliards d'euros de concours de l'État, qui eux-mêmes ne représentent qu'une partie des prêts de 105 milliards d'euros de transferts financiers de l'État aux collectivités, mais derrière ces chiffres, les nombreux élus locaux que nous rencontrons dans le département nous disent leur malaise, leur inquiétude et leur lassitude inquiétude alors que les collectivités ont subi ces dernières années des baisses significatives de dotation alors qu'elles ont dû digérer d'importantes loi portant réforme territoriale qui ont grandement modifié le paysage institutionnel français le territoire Aspire à un peu de répit dans ce contexte, certaines annonces faites au cours de l'été dernier, annulations de crédits, diminution des emplois aidés, etc, ont suscité au mieux de l'inquiétude, mais le plus souvent abattements ou colère ces inquiétudes sont accrus par certains articles de la loi de programmation et de la première partie de ce projet de loi de finances. Règle d'or renforcée et contractualisation aux contours flous avec les collectivités les plus importantes. Si on peut se réjouir de l'abandon d'une logique de baisse mécanique des dotations pour une approche plus partenariale, les modalités de la contractualisation censé s'y substituer, interroges, même si le président de la République a un peu rassuré jeudi dernier en précisant, devant les maires de France, que plus de 99 pourcent des communes n'étaient pas visés. Dans la même veine, je dirai un mot : la disparition progressive de la taxe d'habitation pour 4 Français sur 5 disparition qui n'en doutons pas, sera rétabli à l'Assemblée. Engagement de campagne du président de la République elle satisfait les contribuables qui n'auront plus à s'acquitter de cet impôt inique, du fait notamment de l'obsolescence des valeurs locatives et d'injustifiables disparités. Elle a aussi suscité la crainte légitime dans nos territoires, malgré la promesse d'une compensation intégrale, sous la forme d'un dégrèvement. Pour avoir, comme beaucoup dans cette assemblée, une expérience d'élu, je me souviens de précédents où l'État est progressivement passé d'dégrèvements une compensation avant dans un 3ème temps de rogner patiemment et régulièrement cette dernière. à cet égard je pourrais mentionner la baisse de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, notamment pour les communes, contrairement aux engagements pris par l'État. Mais le président de la République s'il a reconnu qu'il a lui-même reconnu, devant les maires réunis en congrès que l'été n'a pas été à la hauteur de ses engagements à tracer une voie ambitieuse en matière de finances locales. Dans ce cadre, le présent PLF ne serait que la première étape d'une refonte globale de la fiscalité locale, donnons-lui le crédit de s'attaquer à une réforme d'ampleur et trop de fois reporté, il trouvera chez les membres du RDSE des parlementaires exigeant vigilants et soucieux de renforcer la justice et l'autonomie financière et fiscale des collectivités. En attendant cette réforme d'envergure, il nous revient d'examiner les crédits de cette mission. Soulignant tout d'abord, la progression de 95 millions d'euros la DGF qui permet d'augmenter les dotations de péréquation verticale. La déçu et la DSR s'accroissent ainsi de 90 millions d'euros chacune, auxquels il faut ajouter 10 millions d'euros d'augmentation de la dotation péréquation des départements. Les incitations qui sont un des éléments du succès des communes nouvelles ont été prorogés et même renforcé à l'Assemblée, notre groupe proposera d'aller encore plus loin pour encourager les communes qui se lance volontairement dans ces fusions. Les principaux mécanismes de péréquation horizontales, le flic et le Fonds solidarité des communes de la région d'Île-de-France sont quant à eux, maintenus à leur niveau de 2017. Au rang des satisfactions, évoquant l'automatisation du FC TVA prévue à l'article 58, tant sa gestion actuelle est à la fois complexe, illisible et archaïque. Parmi les concours financiers retracée dans le programme 119 la des et gelé en autorisations d'engagement dans le texte initial mais progresse après l'adjonction des 50 millions d'euros, d'une part de l'ancienne réserve parlementaire à cet égard, notre groupe proposera d'améliorer le fonctionnement de la commission départementale chargée de donner un avis sur certains projets retenus par le préfet. Les autres dotations sont également gelés, c'est le cas de la dotation politique de la ville, qui voit la liste des communes éligibles s'élargir, mais aussi la DGT des communes, des départements et des régions, maintenu au même niveau depuis 2009. S'agissant de la décile, si l'on peut se réjouir de son inscription dans le code général des collectivités territoriales, sa pérennisation à son niveau de 2017 dans le programme 119 ne doit pas occulter tous programmes confondus, une diminution des crédits entre 2017 et 2018. Cette évolution aura des répercussions notamment s'agissant du financement des contrats de ruralité, madame la ministre pourrait sans doute nous apporter des éléments sur le financement de ces contrats en 2018. En conclusion, les sénateurs du groupe RDSE seront particulièrement attentifs aux débats qui auront lieu et au sort réservé à leurs amendements en en leur attachement au principe de la limite, administrations et d'autonomie des collectivités, nous serons évidemment réceptifs aux gage de confiance et à la nécessité d'une ligne directrice claire à moyen terme, les élus locaux et nationaux, ont besoin de cohérence lisibilité nous prendrons d'autres décisions, en conséquence, je vous remercie.

présente une façade de stabilité globale en ce qui concerne les ressources de fonctionnement de nos collectivités, on peut affiner la discussion sur les chiffres derrière la virgule, mais enfin l'engagement pris par le président de la République, dès le début de sa campagne, de ne pas agir sur le montant des dotations pour conduire les collectivités à une politique de dépenses retenu cet engagement est tenu et même lorsqu'il y a discussion le retour aux résultats dans 18 mois d'ici lorsqu'on observera les comptes administratifs des collectivités locales fera justice des débats. Mais nous voyons tous que cette stabilité n'est que l'avant- propos d'un projet de transformation. Si j'essaye de. Me remémorer l'ensemble des propos qui sont tenus dans cette assemblée depuis longtemps quant au caractère abîmée, dégradée, devenu trop complexe et illisible du schéma financier des collectivités territoriales, il me semble que cette transformation est reconnu souhaitable pratiquement sur tous les bancs. Simplement, la phrase d'après est déjà un peu plus difficile à écrire, parce qu'ils font après affirmer comment. En tout cas, donc le choix qui est fait et que notre groupe approuve, c'est que les dotations soient préservés mais ça ouvre le débat de savoir jusqu'à quel point elles pourront soutenir un effort de solidarité, ce qui est leur mission, puisque si on conserve la masse mais qu'on fait de la redistribution interne évidemment l'objectif de stabilité de sécurisation des ressources. Et tout de suite touché ce qui nous conduira à me semble-t-il, au-delà des proclamations un peu sonore adopter un schéma d'évolution de la DGF très progressif et allant vers la simplicité, en tirant les leçons de la tentative avortée de la précédente réforme, nous avons convenu entre tous ceux qui participent à la discussion que la redéfinition globale des bases de la DGF se heurter à des obstacles très difficilement franchissables je suis modeste ensuite le 2ème élément de cette transformation. Va être la tentative d'une gestion concertée et responsable du niveau de la dépense locale de fonctionnement. Ceci est une nouveauté pour la France et au contraire une généralité dans l'Union européenne, avec laquelle nous partageons une monnaie commune qui nous crée des obligations auxquelles la France a souscrit de longue date en montrant une difficulté persistante à respecter les 10 engagements. La modération observée sur 2014, 2016 et qui sera très probablement vérifier à nouveau canton n'aura des comptes 2017 montre que cette gestion responsable est possible l'état la portée des gestionnaires locaux, qui sont de toute façon très attention à leurs dépenses et qui ont de plus en plus une vision prospective et ajoutons puisque je ne parle ici que du fonctionnement que si nous sommes capables de. Continuer à contenir l'évolution de nous dépenses locales autour du niveau de l'inflation, si les dépenses si les recettes présente un minimum de dynamique, ce qui est plus facile en période de croissance, ça veut dire que notre marge d'autofinancement, la marge d'autofinancement de nos collectivités auraient vocation à augmenter, ce qui est me semble-t-il souhaitable pour tout le monde. Il reste que le dispositif de contractualisation, je ne vais pas le détailler ici, je n'ai pas le temps, va faire l'objet encore de concertation à la conférence des territoires et puis surtout, d'un débat législatif au cours de la première quinzaine du mois de décembre. La recommandation que fera la mission que je ne d'animer avec le préfet mur sera, que ce soit une première phase et que, à l'horizon 2020 lorsqu'on aura une année complète d'observation, on fasse probablement quelques améliorations quelques-uns à ce dispositif de gestion partagés et concertés. Mais le sujet qui ouvre encore plus de perspective, c'est évidemment la demande qui nous est faite par l'exécutif, là aussi, à partir d'une prise de position claire du président de la République d'engager une rue, une transformation de la fiscalité locale et très vite. Nous allons nous placer devant une bifurcation. Qui est à la disparition d'une recette d'une vingtaine de milliards d'euros, même 23 si on compte tous qui est la taxe d'habitation est-ce que l'objectif. Et de partir sur la création d'une nouvelle imposition locale qui rempliraient mieux les objectifs d'équité que la de, de, de partage, la contribution que la taxe d'habitation. Avec, du coup, le caractère d'une imposition locale autonome et donc un pouvoir de tous. Mais avec. Le petit inconvénient vis-à-vis de la grande majorité des citoyens de dire on a supprimer un impôt, mais on a une bonne idée, on vous en propose un autre. l'autre branche de l'alternative, c'est évidemment une part garantie d'imposition national ayant une dynamique. Ce soir, à se présenter au cours des 6 mois qui viennent. Inutile de dire que les propositions de tous, proposition réfléchi et un peu chiffres sont bienvenues. Et que le moment des récriminations et des protestations évidemment toute sa légitimité mais que l'ouverture vers un avenir équilibré et équitable de partage des charges de fonctionnement du collectivités locales est un débat auquel normalement personne est légitime à ce esquive. Et ceci, je reprends le propos du rapporteur de la commission des lois à l'instant, nous amènera nécessairement à un débat bienvenue et intense sur la conception de l'autonomie nancier des collectivités territoriales, parce que dans le paysage d'inégalités de ressources et d'inégalités de pente économique. De beaucoup de nos territoires, non seulement entre les territoires ruraux certains territoires urbains, mais à l'intérieur des territoires, nous rencontrerons rapidement la vérité inconfortable. Qui est que le maximum d'autonomie et de diversité de ressources locales. Et forcément, producteur du maximum d'inégalités et de différence de chance, c'est ce que je fais Monsieur le Président, il me semble que c'est un choix que personne ne pourra éluder. Merci, merci, je vous ai je joueur rappelé à l'ordre un petit peu tard donc, la parole est à monsieur Pierre Yves Collombat. Monsieur le Président, Madame la Ministre Monsieur a collègues comme on le sait, la mission relations avec les collectivités territoriales 3 milliards

ces crédits ne représentent que 3,8 pourcent du total des transferts de l'État aux collectivités pour reprendre le langage convenu de la LOLF transferts de l'État qui augmente de 1,2 pourcent et l'année prochaine, sur un total de 100 1 milliard 398. Finalement pas trop mauvais millésime pour les collectivités, serait-on tenté de dire ce que le gouvernement ne se prive d'ailleurs pas de faire,

Comme l'a fait remarquer en commission notre rapporteur pour avis, il s'agit là d'une technique de camouflage efficace de la baisse des concours financiers réels de l'État derrière une apparence une un écart de plus de 3 milliards d'euros et 5 pourcent d'ici la fin du quinquennat sauf aussi que les aides financières provenant traditionnellement d'autres ministères et d'autres organismes baissant le résultat final, final risque encore d'être moins brillant intérieure, on l'a dit, suppression de la dotation parlementaire, ministère du Travail, moins 1 milliard globalement sur les contrats aidés, tous ne concerne pas les collectivités, mais quand même une bonne partie, agence de l'eau apparemment la ponction l'année prochaine sera de de 400 millions la liste n'est pas exhaustive, d'ailleurs, comme dit sobrement l'annexe du projet de loi de finances consacré à cette question, l'évolution des subventions des ministères en faveur des collectivités Thériault territoriale, je cite, est difficilement prévisible mais je avoue le principal sujet d'émerveillement pour moi, c'est que l'on puisse continuer à présenter à l'opinion comme des transferts financiers de l'État aux collectivités, donc comme des aides de l'État aux collectivités des compensations incomplète d'ailleurs de transferts de compétences et de charges, notamment à l'occasion des vagues de décentralisation des atténuation des effets pervers de décisions fiscales favorables à telle ou telle catégorie de contribuables mais pénalisante pour les collectivités, la contrepartie âprement discuté de services rendus, dernière en date, les titres sécurisés et bien d'autres choses du même acabit, qui se souvient aujourd'hui que la DGF fossilisé depuis longtemps, a pour origine des taxes locales sur les échanges commerciaux remplacé par les transferts de la taxe sur les salaires, elles-mêmes, même certains s'en souviennent remplacé par verre RTS Rob versement représentatifs de la taxe sur les salaires et puis qu'est devenue la DGF qu'est-ce que le FC TVA sinon le remboursement partiel et souvent avec retard de la TVA qui grève l'investissement des collectivités, on pourrait aussi évoquer le caractère dérisoire de la contribution de l'État au financement des SDIS, dont la direction opérationnelle appartient au préfet, drôle de compétence partagée entre ceux qui dirigent et ceux qui paient quand on fait l'addition, on constate que les transferts financiers de l'État aux collectivités, si l'on entend par là des All réel est plus proche de 30 milliards que 200 milliards, je suis preneur Madame la Ministre de chiffres qui seraient des chiffres officiels mais on nous les a jamais fourni et montrerait encore l'écart qu'il y a entre les apparences et la réalité des transferts financiers de l'État aux collectivités si j'insiste sur ce qui pourrait passer pour une simple affaire de convention, c'est que ce camouflage permet de justifier aux yeux des Français et les médias ne s'en prive pas l'embrigadement des collectivités territoriales dans la croisade contre les déficits publics dont elles ne sont en rien responsables, quoi de plus léger légitime si légitimement elle bénéficiait de 100 milliards d'aides de l'État. La créativité d'ailleurs du gouvernement n'étant jamais prise en défaut, cela permet aujourd'hui de justifier qu'on encadre leurs dépenses de fonctionnement. 1,2 pourcent dans la version du gouvernement initial 1,9 pourcent si j'ai j'avoue avoir un peu de mal à comprendre comment on pourra ainsi réduire signatures significativement l'endettement public étant donné que les sections de fonctionnement qui représentent quelque 80 pourcent des Budgets des collectivités territoriales, étant donné que la dette des collectivités ne représente pas plus de 10 pourcent de l'endettement public, comment on va pouvoir arriver au bout, le seul résultat auquel on va arriver, c'est que on baissera fera baisser encore l'investissement et donc des collectivités, qui représentent 70 pourcent de l'investissement et donc on renforcera la stagnation économique et le chômage, pas du tout, nous dit le 1er ministre. Réduire les dépenses de fonctionnement permettra d'augmenter l'autofinancement, tout en préservant l'investissement sur le papier, ça me fait, ça n'est pas impossible mais dans la réalité avec des collectivités qui sont ponctionnés depuis 10 ans, je pense que c'est hautement improbable. Le plus piquant de l'affaire, c'est que l'on demande aux collectivités territoriales de ce 2 endetté de 67 milliards d'euros d'ici la fin du quinquennat alors que l'État s'endette Raluy de 223 milliards d'euros à s'en tenir aux chiffres fournis par le gouvernement, le résultat serait une baisse de l'endettement public de 5 points de PIB en 6 ans, la dette publique, actuel représentant 96,8 pourcent du PIB, il faudra donc plus de 36 heures de plus de 36 ans pour atteindre la barre des 60 pourcent un peu plus si, entre-temps, les collectivités territoriales mettent la clé sous la porte, vous aurez donc compris que notre groupe ne votera pas les crédits de cette mission. Merci, la parole est à madame Françoise guette-t-elle pour 8 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le président de la commission, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, les collectivités territoriales sortent épuisés du traitement que l'État leur a infligé de manière autoritaire, ces 3 dernières années, elles ont en effet subi un chamboule-tout institutionnel un peu brouillon, une baisse continue et non négociée de leur dotation quand l'État était incapable de s'imposer à lui-même la frugalité qu'il exigeait des collectivités un transfert de charges non ou mal compensée et une augmentation des dépenses obligatoires, je veux parler du jour de carence des rythmes scolaires et des dépenses sociales pour le département et de la voracité normative aussi doit-on souligne avec satisfaction certains éléments proposés dans ce père, je citerai principalement le maintien du niveau de la DGF pour 2018, la diminution de certaines dépenses obligatoires jour de carence maintien du fonds de soutien aux communes, suite à la liberté donnée sur les rythmes scolaires et mais je le souhaite, d'une réforme de la fiscalité locale avec la TVA des régions, même si celle-ci a suscité quelques questions également le renforcement du soutien à la création de communes nouvelles avec un principe de stabilité de DGF une hausse du plafond et la majoration de 5 pourcent de la dotation forfaitaire, toutefois, Madame la Ministre, cette majoration est très minime quand on sait que la création de communes nouvelles s'achèvera au 1er janvier 2019 en raison des échéances municipales en 2020 et je regrette la faiblesse de l'encouragement alors que les communes nouvelles sont une dépense d'investissement pour l'avenir, répondant au double besoin de proximité, d'efficacité et à la consolidation de centralité certes, mes chers collègues, peut-on continuer de donner plus à des communes qui fusionnent au détriment des autres puisqu'il s'agit d'une enveloppe fermée, c'est pourquoi je proposerai afin de ne pas pénaliser l'enveloppe de la DGF des communes et des intercommunalités particulièrement contrainte de créer un fonds dédié aux communes nouvelles, cela a été fait pour les métropoles et les communautés d'agglomération, le coût des communes nouvelles est très faible, il a été de 2 millions en 2017. Contre 70 millions pour les communautés d'agglomération, la difficile Madame la ministre aurait pu constituer un motif de grande satisfaction car la hausse important affichée en autorisations d'engagement si elles n'étaient pas le fruit d'une habileté de présentation, car il faut en convenir, la hausse est avant tout liée à un changement de périmètre, en effet, si l'on neutralise ces effets de périmètre les autorisations d'engagement diminueraient de 255 millions d'euros, soit une baisse de 29 pourcent je note avec satisfaction qu'en compensation de feu la réserve parlementaire nos collègues députés ont souhaité réaffecter une enveloppe de 50 millions d'euros pour les communes et interco engagé dans un projet de modernisation je félicite notre rapporteur pour la création de la commission départementale des investissements locaux qui permettra aux élus locaux et nationaux d'être partie prenante dans l'attribution de la destinée de la de Je souhaiterais maintenant Madame la ministre et quelques exemples évoquer la question de la compensation du transfert de charge, avec notamment l'augmentation de la dotation forfaitaire relatives à la délivrance des titres sécurisés, je veux parler des passeports et des cartes nationales la hausse qui figure dans le budget n'est hélas pas lié à une revalorisation de la compensation pour les communes déjà équipés, mais elle est liée à la seule augmentation du nombre de communes accueillant un dispositif de quid du Pacs, les maires se sont vu attribuer ses compétences d'état civil précédemment exercé par les tribunaux d'instance exercée par les maires, dans le cas de leur qualité d'agents de l'État, les compétences transférées nouveau selon la jurisprudence du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, pas droit à compensation, or l'article 31 du projet de décret prévoit que le transfert des données numériques et des dossiers papier détenus par les grèves des tribunaux d'instance aux officiers d'état civil des communes siège dès lors les communes siège de tribunaux devront traiter le Pacs pour l'ensemble des communes, ne croyez-vous pas, Madame la Ministre, que cette charge supplémentaire mérite une indemnisation, telle que proposée par un amendement sénatorial, Madame la Ministre, la mission relations avec les collectivités territoriales ne correspond qu'à 3,6 des transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales, donc vous comprendrez la nécessité d'élargir mon propos et je voudrais parler de la réforme de la taxe d'habitation sur l'injustice de la taxe d'habitation est exact, pourquoi ne les votons pas pour le foncier bâti le Sénat représentant des territoires, vous comprendrez madame la Ministre, peut difficilement accepter en l'état, la disparition de de ressources majeure sans aucune information information et précision préalable sur la nécessaire refonte de la fiscalité locale, que le président de la République a également appelé de ses voeux, les élus ont besoin un besoin impérieux de stabilité et de prévisibilité, ils doivent comme d'chute du chemin pour définir le meilleur trajet à emprunter, ne croyez-vous pas, Madame la Ministre, que cette absence de visibilité présentent un risque de ralentissement de la politique d'investissement des collectivités si nécessaire à l'économie locale, enfin, Madame la Ministre, vous conviendrez que la suppression de la taxe d'habitation, confort de l'inégalité entre communes, car ce sont les communes les plus pauvres qui seront les plus lésés, on peut effectivement préféré comme vous le proposez de manière en soit pertinente la contractualisation financière entre l'État et les collectivités une base universelle et autoritaire des dotations mais toutefois vous conviendrez qu'il est difficile à ce stade d'apprécier le mécanisme de contractualisation, il convient d'en savoir plus sur les conclusions de la mission préparatoire confié à notre éminent collègue Alain Richard et Dominique Bur et les suites qui seront données pour ma part, je m'interroge sur l'intégration des dépenses obligatoires, dont l'objectif de diminution des dépenses de fonctionnement dépenses obligatoires qui, par nature, échappe à l'initiative des collectivités, je veux parler de la revalorisation du point d'indice du RSA enfin un contrat est un pacte défini et négocié entre 2 partenaires alors sera-t-il impact forcé avec une règle d'or renforcée, c'est un partenaire refuse de signer, vous avez compris, Madame la Ministre, le groupe centriste, salut les éléments positifs de ce projet de loi de finances et la fin d'une politique autoritaire de rabot budgétaire et de transferts de charges non compensés et en même temps ça se dit beaucoup aujourd'hui, et là je le crois profondément, Madame la Ministre, et en même temps avec les collectivités, que le Sénat représente nous aspirons à ce que soit engagée une vraie réforme des finances locales avant toute suppression de la taxe d'habitation, une réforme basée sur l'adéquation des ressources avec des charges transférées le lien entre les compétences et les ressources mais aussi le lien entre le contribuable local et le financement des services publics et la garantie de la libre administration des collectivités, vous l'avez compris, Madame la Ministre, la position du groupe centriste est à la fois un encouragement et un avertissement nous serons très vigilants sur la mise en oeuvre du discours du président de la République qui, sur les exigences de nos territoires, aussi le groupe centriste dans sa majorité s'abstiendra-t-il encore une fois, cette abstention est à prendre comme un encouragement et un avertissement : je vous remercie. Merci, Merci, la parole est à monsieur Didier Marie pour 10 minutes. Seul président, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous examinons ce matin dans le cas de la mission, relations avec les collectivités territoriales, l'affectation d'une enveloppe de 3,8 milliards d'euros sur les 104,6 que représentent les concours de l'État aux collectivités, soit 3,6 c'est peu mais c'est un zoom qui permet d'appréhender cette relation en la replaçant dans son contexte. De 2014 à 2017 les collectivités appelées à participer à l'indispensable effort de redressement des comptes publics ont été au rendez-vous en 2014, 2015 et 2016, leurs dépenses ont diminué respectivement de 0 1,1 pourcent et 0 8 alors que l'prévoyait une augmentation de 1,2 0 5 et 1,9 soit au final 21 milliards d'euros d'économies 12 de plus que prévu par la précédente loi de programmation des finances publiques. Ainsi, la réduction du déficit public, a été porté à hauteur de 60 pourcent par les administrations publiques locales alors qu'elle ne représentait que 20 pourcent des dépenses cet effort mené de manière responsable, a atteint ses limites et pèse aujourd'hui sur les dépenses d'investissement qui ont baissé en 2016, 2 3 pourcent alors que la croissance repart, que les comptes publics s'améliore, que le déficit ne devrait plus dépasser les 3 c'est encore aux collectivités que le gouvernement demande de faire des efforts, c'est à la fois injuste et inefficace, injuste, car elles ont tenu leurs engagements et que bon nombres d'entre elles pour continuer de maîtriser, voire de baisser leurs dépenses devront remettre en cause non plus des dépenses superfétatoires, mais des services rendus à la population, la plupart des collectivités, excusez-moi l'expression, atteint l'os, il n'y a plus rien à gratter. Inefficace car au final, la variable d'ajustement sera leur capacité d'autofinancement et donc d'investissement, ce qui ne sera pas sans impact sur l'économie, le secteur du BTP en particulier et donc sur l'emploi. Si l'on peut souscrire à la fixation d'un objectif d'évolution des dépenses des collectivités, la progression en valeur et par à 1,2 pourcent inflation comprise, est intenable à ce sujet, le rapporteur général de la commission des finances, a démontré que l'évolution tendancielle des dépenses retenues étaient largement sous-estimé, excluant les efforts déjà réalisés et ne prenant pas en compte la non-indexation sur l'inflation des rémunérations des fonctionnaires territoriaux ainsi l'objectif n'est pas de 13 milliards d'euros d'économies, mais de 21 milliards d'euros, ce qui équivaut, soyons sont assurés d'une baisse nette des dépenses de fonctionnement du collectivités territoriales. De même, le plafonnement des ratios d'endettement dit règle d'or renforcée pénalisera les investissements, prenons l'exemple d'un département peu endettés en 2017 qui décide d'investir massivement en 2018 et en 2019 dans le déploiement de la fibre optique, prévoyant d'amortir cet investissement par l'intermédiaire d'une redevance sur 30 ans.

quant à ce que le gouvernement appelle pudiquement le mécanisme de correction en cas d'écart entre les objectifs fixés, la réalisation, c'est particulièrement vécu comme déplaisant et infantilisant par les élus locaux. Ceux-ci sont responsables et il ne semble pas judicieux de brandir la règle pour leur taper sur les doigts d'autant que le maître en l'espèce, l'État est loin d'être irréprochable. Madame la Ministre des élus sont inquiets et leçon de cette volonté d'aller trop loin dans l'obligation que vous leur faites de réaliser toujours plus d'économies et de renoncer aux politiques publiques, ils ont mis en place au bénéfice de leur population, ils le sont car une part des économies se fera sur le dos des agents de la fonction publique territoriale qui verront leur point là dit je et le jour de carence rétablie. Ils le sont parce qu'ils ne partagent pas le pari du gouvernement sur la baisse des dépenses sociales en particulier celles des départements pour le qui pourrait bien d'être démenti par les chiffres du chômage toujours à la hausse. Ils sont inquiets, Madame la Ministre, de cette suppression progressive de la taxe d'habitation bienvenue pour les contribuables, mais qui ne résout d'aucune façon les inégalités entre ceux-ci ni celle entre les communes, mais qui disent en un peu plus ce lien civique entre l'impôt et le citoyen. Le président de la public nous promet une grande réforme de la fiscalité locale en 2020. Soit, mais qui peut croire que l'or, on viendra sur l'effacement de la contribution des ménages sous quelque forme que ce soit la remise en cause de la taxe d'habitation, certes injuste et inefficace, aurait mérité, une vraie réforme de la fiscalité, j'en viens aux quelques articles de cette mission qui nous occupe ce matin, on ne peut Madame la Ministre, que constater et regretter que les dotations décentralisation versées à la suite de transfert ou de maintien, de compétence, gelé depuis 2009 le soit encore et poursuivent leur lente érosion. Si la pérennisation de la dotation de soutien la local est une bonne décision, il convient tout de même d'en relativiser la portée lorsque l'on constate que l'ensemble des dotations d'investissement subissent une coupe sévère en autorisations d'engagement due pour l'essentiel à la non-reconduction des fonds de soutien aux régions et à la suppression de la réserve parlementaire je regrette par ailleurs l'intégration de la dotation de compensation de la taxe professionnelle du bloc communal au variable d'ajustement qui baisse de 8 pourcent et qui va pénaliser les territoires anciennement industrialisés, décision qui suit l'intégration en 2000 17 du fonds départemental de péréquation n'a taxe professionnelle au même variable d'ajustement qui, lui, baisse de 17 pourcent cette année, ce qui n'est pas acceptable pour les communes de défavorisées qui en bénéficient, dans mon département, la Seine-Maritime, dans laquelle vous venez samedi prochain à l'occasion de l'assemblée générale des maires, ce fonds est une composante essentielle des ressources de bon nombre de communes rurales défavorisées pour elle, cette baisse met en danger leur équilibre budgétaire car peut représenter jusqu'à 20 pourcent de leurs recettes de fonctionnement, vous ne manquerez pas j'en suis sûre d'être interrogé sur ce problème. quant elle, après avoir progressé en 2015, 2016 et 2017 ne continue pas sa progression au même rythme, tout comme les contrats de ruralité seulement doté de 45 millions d'euros, montant bien inférieur aux besoins

Ainsi, madame la ministre, la défiance l'emporte sur le pacte de confiance, la liberté l'administration des collectivités et progressivement remis en cause au bénéfice d'une recentralisation illustrées par la distribution à la main, des préfets, des dotations d'investissement à nos collectivités. Nous apporterons dans la discussion des propositions d'amélioration comme la constitution d'une commission unique pour les investissements locaux, la gestion de ceux-ci au niveau départemental, en présence de parlementaires ainsi que une proposition d'abaissement du seuil de de l'examen de ces projets à 50000 euros, mais sur le fond, nous ne pouvons souscrire à vos propositions qui relèvent au final d'un affaiblissement des collectivités territoriales et de leurs capacités d'investissement pour merci. Merci, la parole est à monsieur Philippe Dallier pour 5 minutes. Monsieur le président, madame la ministre, le président de la commission des finances, messieurs les rapporteurs, chers collègues, tous les maires et plus généralement tous les élus attendaient beaucoup du discours de Monsieur, le président de la République devant le 100ème congrès de l'Association des maires de France, ont-ils été rassuré ses élus, je crois que la réponse ne soit assez généralement non pourquoi, tout simplement parce qu'il n'y voient pas beaucoup, beaucoup, beaucoup plus claire après qu'avant, certes, le président de la République a tenté de 2 miné le terrain du projet d'exonération de la taxe d'habitation pour 80 pourcent des Français et de l'encadrement de la hausse des dépenses des plus grandes collectivités territoriales afin de trouver les 13 milliards d'euros d'économies retenu comme objectif par le gouvernement, mais pour autant, les décisions le détail de ces mesures sont renvoyées à plus tard ainsi au moment d'examiner les crédits de cette mission, nous devons nous contenter de la promesse de stabilisation de la DGF jusqu'en 2022, et de celle d'un Big bang de la fiscalité locale en 2020 afin de sortir de l'épineuse question de la taxe d'habitation concernant la DGF après 4 années de baisse très importante qui ont conduit beaucoup de nos collectivités aux limites du supportable l'engagement du gouvernement ne rassurent pas complètement rappelons d'abord que cette promesse ne se traduira pas par une stabilité des dotations de l'État pour toutes les collectivités, puisque dès 2018 certaines continueront à voir leur dotation baisser, en effet, la progression de la DGF pour les collectivités, gagnant la population ou par exemple les bonifications accordées en cas de création de communes nouvelles se font au sein d'une enveloppe fermée cette progression pour les uns, et donc une baisse pour les autres, mais il y a aussi la progression des dotations de péréquation, ce sera le cas de la DSR et la DSU en 2018 qui jouera sur les variables d'ajustement desserte épais ou la dotation de compensation des exonérations de taxes foncières continueront à baisser pour les communes et les EPCI un mot particulier sur la desserte pour rappeler, elle est l'archétype des dotations à leur création compenser une perte de recettes pour nos collectivités et qui au fil du temps s'étiole rompant la promesse de l'État, c'est d'autant plus injuste que cette dotation bénéficiaient principalement aux collectivités ayant subi une perte de base d'imposition et donc de produits au moment de la réforme de la taxe professionnelle et ce sont en général des collectivités au passé industriel et aux population souvent modeste en première partie de ce PLF le ministre alors au banc, Olivier Dussopt a laissé entendre que le gouvernement réfléchissait à une modification des règles de calcul de la baisse de cette variable d'ajustement afin de moins pénaliser ces collectivités incident que nous pourrions bientôt avoir pour cette variable d'ajustement, la prise en compte d'une forme de péréquation, ça va me semblait extrêmement compliqué, mais il y a aussi les changements fréquents des règles de calcul des dotations de péréquation c'est encore le cas cette année avec la DSU après la décristallisation de l'année dernière et cette année encore, je constate que beaucoup de nos collègues ont déposé des amendements proposant de changer à nouveau les règles de calcul du pic, chacun essaie essayant disons le très clairement de tirer la couverture à lui mais tout cela se fait forcément au détriment de tous les autres, alors je crois mes chers collègues, que nous ne pouvons pas continuer ainsi, non seulement beaucoup d'élus locaux ne verront pas se concrétiser la promesse de stabilité de la DGF du fait des décisions du gouvernement mais aussi de notre propre responsabilité, je crois qu'il aurait été bien plus sage de décréter un moratoire et je rejoins mon collègue Claude rénal sur les règles de calcul, ainsi que sur les montants de chacune des dotations dans l'attente d'une véritable réforme de la DGF et de l'ensemble de ces dotations de péréquation car chacun voit bien que notre système est à bout de souffle le bateau prend l'eau de toutes parts et en voulant combler une brèche, on finit toujours par en ouvrir une autre, madame la ministre sait bien que c'est un chantier compliqué mais vous devez l'ouvrir la commission des finances du Sénat a déjà beaucoup travaillé, même avec l'Assemblée nationale l'an dernier, que deviendra ce travail, c'est toute la question, voilà la milice, nous avons besoin d'une réponse et puis, il y a l'autre chantier, celui de la fiscalité locale, là aussi je trouve regrettable que nous ne l'avions pas plus vite, certes il y a la promesse électorale du candidat Emmanuel Macron de supprimés en 3 ans, la taxe d'habitation pour 80 pourcent des Français, mais nous savons tous, et lui aussi va ailleurs le sait que pour des raisons constitutionnelles cela se terminera par la suppression complète de cette taxe, il a d'ailleurs laissé entendre lors du congrès des maires, mais alors, par quoi la remplacer par la totalité de la taxe foncière attribuée aux communes cela couperait le lien entre une grande partie des habitants, ce qui ne sont pas propriétaires et le financement des services publics locaux et puis surtout, cette taxe foncière sera-t-elle toujours assis sur des valeurs locatives obsolètes, que nous n'aurions pas eu le courage de le réviser madame la Mini, je crois que ça n'est pas possible autre solution : remplacer la TH par un autre impôt qui préserverait le lien avec les habitants, d'une part d'impôt sur le revenu, pourquoi pas, mais il y aura alors l'inconvénient politique parce qu'en 2020, certains qui auraient été exonéré complètement de taxe d'habitation, pourrait se trouver éligibles à cette ont autant que vous avez là un autre problème politique, voyez-vous, je suis prévenant à l'égard du gouvernement et voilà pourquoi je vous dis, Madame la Ministre, que vous ne pouvez pas attendre 3 ans, il faut aller vers cette grande réforme fiscale et pour terminer, je dirais simplement comme l'un de mes collègues que nos communes, nos départements nos régions, nos Interco ont besoin de visibilité, elle n'est pas là cette visibilité et il est fort à craindre effectivement que ça soit l'investissement public local

monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, chers collègues, il n'est pas anodin de trouver dans le sud de cette mission dédiée aux collectivités territoriales le terme relation cette dernière suppose de partis qui, si elles ne doivent pas toujours s'apprécier sont tenus en revanche de se respecter et de s'entendre cela exclut donc toute velléité domination de l'une sur l'autre, en un mot, cela nécessite de la confiance réciproque, or force est de constater qu'entre l'État et les collectivités, le courant ne passe plus la défiance de chaque côté, règnent en maître, j'étais maire, je sais que ces élus dans une large majorité, bénévoles et qui ne comptent pas leurs heures sont chaque jour confrontés à des choix impossibles enserré entre le marteau et l'oncle entre nos concitoyens qui attendent beaucoup de ce qu'il considère comme le 1er représentant l'autorité ou une dernière protection et l'État qui leur demande toujours plus, en leur accordant toujours moins de moyens, j'ai été président du conseil départemental, je sais les défis auxquels cette collectivité confronté baisse des dotations, explosion des dépenses sociales dont le RSA qui ne sont pas compensés par l'État et qui, quant à lui, paradoxalement, est en charge de la lutte contre le chômage, prise en charge exponentiel des mineurs étrangers isolés, alors que le sujet des flux migratoires, relève, celle de l'État, ainsi les départements assume ce que l'État veut ignorer, j'ai été longtemps député avant d'être un nouveau sénateur je sais l'exercice convenu et l'outil de communication politique que le budget représente pour tout nouveau gouvernement mais je vous invite ici à en sortir ce 1er budget doit être pour vous l'occasion d'envoyer un message fort à tous ces élus qui, sur le terrain se battent avec les moyens limités dont il dispose pour parler budget après budget, un État qui est aux abonnés absents, lorsqu'il s'agit de mettre la main au portefeuille, car à l'inverse, pour imposer des contraintes transférer des compétences ou créer de nouvelles charges. L'inventivité de certains comptables à Paris attend des sommets, bien loin des réalités de l'implication concrète de ces mesures sur la vie quotidienne de nos compatriotes, ce 1er budget doit être l'occasion de revenir sur des signaux particulièrement hostile à l'égard des collectivités, que dire de la suppression brutale des contrats aidés, que dire de la suppression de la réserve parlementaire et de sa transformation en un dispositif recentraliser et inégalitaire, que dire de la baisse des APL qui a un impact très important pour les collectivités, que dire des 300 millions d'euros de crédit en moins, notamment de la DE Terre dès juillet avant même de les avoir rencontré une relation, mais ce n'est pas décidée et imposée, pourtant, ce 1er budget ressemble à s'y méprendre à cela pour 3 raisons les objectifs d'économie assigné aux collectivités locales, tout d'abord elle ne prennent en aucune manière compte des efforts déjà réalisés consenties par elle, qui ont permis à la France de respecter ses engagements européens, vous promettez le bâton aux collectivités qui ne respecteraient pas une augmentation inférieure à 1,2 pourcent en valeur des dépenses de fonctionnement sans pour autant proposer la moindre carotte. à titre d'exemple, en 2 ans, le conseil départemental que j'ai eu l'honneur de présider dans l'Oise, jusqu'en septembre, a réalisé plus de 80 millions d'euros d'économies sur les 250 millions d'euros de budget de fonctionnement hors dépenses contraintes et cela sans augmenter ni les impôts ni la dette et tout en préservant l'investissement, ce n'était pas mon choix, mais une obligation au regard de la situation financière de la collectivité, il est tellement plus facile de dire que tout va bien et de cacher les problèmes sous le matelas, il s'agit d'un effort sans précédent qui implique des choix clairs et assumés en terme de réduction de la masse salariale notamment ainsi demain, demanderez-vous de nouveaux efforts à cette collectivité la stabilité désengagement financier de l'État en trompe l'oeil, ensuite car il s'il faut saluer la quasi-stabilité des crédits notamment le maintien de la DGF au même niveau que l'année précédente, certaines inquiétudes demeurent, je pense à votre volonté d'inclure dans le périmètre des variables d'ajustement, la desserte RTP du bloc communal, ce choix est très contestable, car l'État revient ainsi sur l'engagement pris en 2009 de compenser intégralement les pertes de recettes subie par les collectivités territoriales, en raison de la suppression de la taxe professionnelle. La réforme de la taxe d'habitation, enfin si une réforme de la fiscalité locale peut paraître opportune et souhaitable, pourquoi ne pas prendre le temps de l'envisager dans son ensemble, pourquoi la prendre par le petit bout de la lorgnette car risques constitutionnels importants mis à Paris gains économiques contrasté pour les particuliers, le mécanisme proposé conduit à une perte d'autonomie financière pour les communes et menace leur survie, puisque d'un côté vous leur refusez une recette dynamique et de l'autre vous compenserait à l'image de ce qui a été fait pour la taxe professionnelle, en effet, nous savons tous ici, ceux que compensation par l'État signifie Madame la Ministre, pire cette décision distant toujours davantage le lien entre les Français et l'utilisation de leurs impôts, tout comme leur lisibilité et alimentent le ras-le-bol fiscal en réalité vous demander à d'autres les efforts que vous refusez de faire pour vous-même, Madame la Ministre, vous avez été maire d'une métropole, on ne peut pourtant vous taxer donneront sur cette question, Madame la Ministre, prenez garde, n'a sans doute pas effectivement madame la ministre, les gare à ne pas confondre pas de confiance et une mise sous tutelle, Madame la Ministre, les collectivités locales ne sont pas une variable d'ajustement que l'État peut à loisir ponctionner remodeler une relation exige des partenaires traiter les collectivités territoriales comme telle. Merci, la parole est à monsieur Henri Leroy pour 5 minutes.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je souhaitais attirer votre attention sur la pente dangereuse vers laquelle le gouvernement entend elle nous amener dans cette réforme inavoué de la fiscalité locale, la combinaison du PLF 2018 et le projet de loi de programmation des finances publiques 2018, 2022 promettent un avenir plus qu'incertain pour la décentralisation des décisions des collectivités locales et leur autonomie financière, principe constitutionnel de notre droit, déjà mise à mal par une belle espèce persistante depuis plusieurs années, il y a, responsable locaux s'inquiètent de la diminution de leur marge de manoeuvre en terme d'investissement pour le prochain quinquennat de 2011 à 2016, les Parm brut des 3 échelons des collectivités locales a diminué considérablement du fait du 10 engagements financiers de l'État. Afin de respecter leur mission de service public, les collectivités locales ont dû recourir de façon irrémédiable et responsable à l'emprunt pour continuer à investir, mais alors même que les exigences drastiques de maîtrise des dépenses de fonctionnement sont imposées par les dispositions du PLF 2018 aux collectivités territoriales, le projet de loi de programmation des finances publiques achève le processus d'affaiblissement, en effet, ce projet de loi de programmation les incite affecter le montant total des économies si difficilement réaliser à la réduction de l'empreinte, s'il est parfaitement concevable que les collectivités territoriales et leurs groupements participent au redressement des finances publiques afin que la France respecte ses engagements européens, cela ne doit se faire qu'à juste proportion de leur part de déficit dans ces conditions, comment le passé mouvoir devant les dispositions de la loi de programmation dont cadrer davantage recours à l'emprunt par le principe de la règle d'or renforcée, laquelle pas un mécanisme raccourcissement du remboursement de l'emprunt neutralise toute possibilité d'investissement l'intégralité de économique si j'ai des collectivités locales en matière de dépenses de fonctionnement devraient affecter à la réduction de leur empreinte certes l'objectif imposé de ce dispositif ou collectivités de réduire leurs besoins de financement, mais il est aussi et surtout restrictif de leur libre administration car enfin, si j'ai 2 projets de loi met fin à la baisse brutale des concours financiers de l'État, nous nous devons de déplorer néanmoins une augmentation des dotations d'investissement de l'État, les autorisations d'engagement étant susceptibles de diminuer si l'on neutralise les effets de périmètres, sans parler de la suppression de la taxe d'habitation pour 80 pourcent des foyers, que dire des dotations d'investissement de soutien à l'investissement local qui sont attribués arbitrairement par les préfets, selon les projets locaux sans concertation aucune avec les élus concernés, je tiens a rejoint tous mes collègues, qui voit dans ces pratiques centralisatrice, un manque de transparence, et incidemment fort peu de considération pour idée du terrain que nous sommes. Nous pourrions également évoqué la perte sèche que constitue la suppression de la réserve parlementaire pour pour nombre de petits projets qui ne verront plus le jour, c'est pourquoi j'apporte un soutien appuyé et sans réserve à notre rapporteur, le sénateur Loïc Hervé lorsqu'il propose de créer une commission départementale des investissements locaux dont la compétence porteur étant sur la DSI elle que sur la DOTS, elle aurait pour Avantage d'être composé de tous les échelons locaux car enfin notre rapporteur dans son rapport, mais parfaitement évident, je cite, une reprise en main par l'État, que ni les hauts lieux locaux ni laisser là ne peuvent insectes et le gouvernement consent moins généreusement, qu'il n'y paraît, leur accorder des dotations d'investissement, c'est pourquoi l'amendement s'85 adopté par la commission des lois, qui propose d'intituler cette commission départementale des locaux ne résultera pas tout mais apporte un début de réponse, cette initiative participe à l'impérieuse nécessité de calme et de soigner l'exaspération les sentiments d'abandon et de déconsidération que ressentent aujourd'hui bon nombre d'élus de terrain, nous revendiquons la liberté d'entreprendre et avons besoin de perspectives, par le biais des finances locales, Madame la Ministre, vous étiez vous-même un élu, il n'y a pas si longtemps. vous devez de faire confiance aux élus locaux qui le méritent, vous le savez bien alors redonner leur l'espoir merci. Merci donc la parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur pour 20 Minutes la ministre. Je suis plus près. Bien, monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, nous étudions aujourd'hui la mission RCT, qui porte sur 3 milliards 8 d'euros. Bien entendu, la discussion a été beaucoup plus large, elle a porté sur l'ensemble de la politique financière du début du du gouvernement et des réformes qui sont en cours mais pour réponde à bord à la mission RCT. J'ai noté consciencieusement les baisses que vous m'avez les uns et les autres annoncés, soit de 8 pourcent soit de 12 2 5 de 13 et de 10 D. pourcentage très variable selon les modes de calcul. Si bien que je vais me. Je vais simplement me limiter, si je puis dire à vous dire que. Depuis 2014, les crédits de dotation d'investissement sont passés de 716 millions d'euros. à 1 milliard

donc on peut effectivement trouver des tas de pourcentages mais tout de même, ça fait une augmentation qui est toute même assez significative depuis 2014 est-ce pas et qui montre que, il n'y a pas de baisse de de dotation d'investissement sur ces crédits, à part les dotations des investissements, il y a bien sur les dotations liées à des transferts de compétences dont le montant est dû et figé, c'est-à-dire environ 2 milliards d'euros, voilà pour les chiffres de la mission RCT de façon brute. Je vous remercie tous d'avoir, d'être intervenu avec plus ou moins de confiance pour plus ou moins de défiance par rapport à la politique gouvernementale, je ne vais pas répondre à tous les points, bien évidemment, puisqu'on aura l'occasion au fur à mesure des amendements dit répondre mais je voudrais revenir sur quelques points qui ont été souvent évoquée, la taxe d'habitation la taxe d'habitation, je sais que le Sénat a pris une position, je rappelle simplement que c'était un engagement du président de la République dans sa campagne et qu'il applique son engagement, ce qui finalement n'est pas si mal, entre ce que l'on dit que l'on va faire et ce que l'on fait, c'est déjà ça n'a pas toujours été le cas, je rappelle par ailleurs que sur les bases locatives les bases cadastrales c'est vrai qu'elles n'ont pas été réévalué. évidemment, et on peut pas forcément porté rigueur au gouvernement actuel qui est là depuis 6 mois puisque depuis des années et des années, comme le rappelait un certain nombre d'élus, j'ai été maire pendant 25 ans, je suis encore conseillère municipale et conseillère communautaire, comme la loi le permet et on sait tout ce qu'il y a eu plusieurs tentatives. Et que, elles n'ont pas abouti et je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de d'en partager la responsabilité aussi bien les gouvernements qui se sont succédé, les parlementaires et les élus locaux qui en voyant les évaluations possibles d'évolution des valeurs cadastrales et les répercussions sur les taxes habitation faisait que tout le monde disait ce top pour qu'on arrête la réforme, ça t'es quand même une réalité, donc je crois qu'il faut toujours dire les choses telles qu'elles ont existé, par ailleurs, je rappelle que la volonté du président de la République était aussi de redonner du pouvoir d'achat enfin quatrièmement que certes, j'ai entendu tout ce que vous avez dit, mais que c'est un dégrèvement c'est sur 3 années, et que donc il y a une garantie de ressources réelles sur ces 3 années, et que la la dynamique de la taxe d'habitation et évidemment respectée puisque chaque année, les services fiscaux donne des bases qui évolue avec le nombre de constructions nouvelles et que la liberté de ton et respecter chacun sait que il n'y a pas d'inquiétude, et vous savez sur le produit attendu comme on dit voter dans les communes et que cette réforme peut s'appliquer dès l'année prochaine, mais naturellement, et c'est le 2ème, point sur lequel je voudrais insister, c'est ceci doit se situer dans une perspective que vous avez tous évoqué de réforme de la fiscalité locale évidemment et je remercie tous ceux qui l'ont dit, ils l'ont proposé et qui y réfléchissent déjà et qui travaillent déjà, c'est une des missions confiées à Alain Richard et au préfet sur la réforme de la fiscalité locale et comme il y a dit tout à l'heure, lui-même toute l'et les participations toute idée faisant vivre le débat est la bienvenue, bien évidemment, il y a eu des rapports très intéressés, très intéressants, qui ont été rappelé tout à l'heure par nos collègues, Charles Guené et Claude rénal qui ont été faits avec des comparaisons avec d'autres pays comme l'Italie ou l'Autriche, toutes ces contributions doivent venir enrichir le débat dans le cadre de la conférence nationale des territoires, c'est bien sûr quelque chose auquel tout le monde doit participer et on ne peut pas concevoir cette réforme de la fiscalité locale sans poser le problème aussi de la définition comme Alain Richard l'a dit tout à l'heure qui a été posée par le rapporteur de la commission des lois, c'est-à-dire la définition de l'autonomie fiscale des collectivités territoriales, c'est quelque chose de très important et je je n'ai pas entendu, c'était même une réclamation des régions que d'avoir une part d'un impôt national, qui est la TVA, dire qu'ils avaient perdu leur autonomie fiscale, je crois qu'ils sont heureux de recevoir une part de la TVA Akitani un impôt dynamique et que, au fond, ça leur permettra d'exercer les compétences nouvelles qui sont les leurs, donc c'est un vrai débat et c'est pas la peine de se jeter des choses à la figure, il faut réfléchir, si à chaque niveau de collectivité locale, c'est la même chose ou s'il faut garder des impôts avec un lien local et un taux, c'est une question qui est posée, donc il faut réfléchir et construire pour effectivement. Essayer de construire un un système si je puis dire, un écosystème comme a dit Charles Guené tout à l'heure, nouveau qui doit tenir compte aussi de l'évolution de nos collectivités locales de l'environnement, ambiance des contraintes européennes Alain Richard a rappelé. De manière, j'ai trouvé très concrète et très pédagogique que nous avons une monnaie commune et que c'est parce que nous avons une monnaie commune de nouveau devront être coresponsables, aussi bien l'État à la sécurité sociale, que les collectivités territoriales et les autres pays liés par la même monnaie à ses engagements que nous avons de maintenir bien sûr le niveau d'endettement en-dessous de 3 pourcent du PIB, donc ce sont des chantiers très importants et toute participation, je crois, et bienvenue. Une 3ème chose aussi qui a été souvent évoquée, c'est de dire au fond. Comment dire, l'État ne fait pas confiance aux élus locaux, bon alors ça c'est un leitmotiv, qu'on a entendu tout l'été, voilà alors le président de la République a lui-même reconnu qu'il avait eu des, des prises de de décisions peut-être un peu maladroite et malheureuse autour de l'été ou mal expliqué de façon. Pas assez pédagogique bon, soit, mais quand je vous entends, je pose en tant qu'élu local, comme chacun l'a rappelé la question enfin est-ce que c'était une marque de confiance que de prélever alors traînement sur la DGF ces dernières années, comment dire, ce prélèvement qui, au fond, avec toutes les conséquences que vous avez évoqué était très dur, très rude, sans discernement, c'était quand même quelque chose de très important, là nous passons à une période où on ne prélève plus sur la DGF ou le montant des dotations d'investissements sont globalement maintenu et troisièmement, où on dit on va contractualiser avec les 319 plus grandes collectivités qui représente à peu près 60 pourcent de la dépense publique nationale, bon et les autres, on leur fait confiance, justement en essayant de limiter effectivement la progression des dépenses à 1,2 pourcent c'est-à-dire, au fond, maîtriser la progression de la dépense en ce qui concerne les contrats, bien entendu, pour répondre à plusieurs orateurs, ils seront individualisés par exemple le prêt, l'ancien président du conseil général de l'Oise qui vient de s'exprimer, les efforts qui ont été faits par le conseil général de l'Oise dans les années précédentes, seront pris en compte c'est, c'est évident, la démographie, sera prise en compte. Alors il y a une chose que je vous accorde, c'est je parle toujours d'Alain Richard c'est que Alain Richard et monsieur Bur sont entrain au même rendu. Un 1er rapport qui va être rendue publique lors de la conférence des territoires du 14 décembre on peut même avant très bien et qui va donner au fond comment dire des détails plus avant sur à la fois ces contrats et la manière dont dont on fera le bilan de ces contrats, c'est vrai qu'on construit en même temps si je puis dire, cette qu'on sera contractualisation mais c'est justement une preuve de discussions de souplesse et de discussions avec l'ensemble des élus voilà je, je tiens à le dire de cette manière et je pense qu'on ne peut pas donc parler de défiance envers les collectivités territoriales et je le dis en pensant que la période précédente, me semblait beaucoup plus rude, alors ce n'est pas facile, c'est jamais facile pour quelque gouvernement que ce soit s'aurait été une autre majorité au pouvoir, je pense que ça aurait été difficile aussi, donc il faut. Essayer de sortir de cette idée. Il y a au fond. Des solutions qui sont évidentes : essayer donc de construire ensemble des réponses à la situation de notre pays en tout cas. Je voulais vous dire au cours de. Des différents amendements qu'il vous qui vont être présentés, je répondrai certain nombre de points peut-être dira à Philippe Dallier,

profiter de cette période. Qui s'annonce pour faire la réforme de la de la fiscalité locale, bien évidemment, je voudrais peut-être dire une chose aussi ce qu'on a beaucoup parlé de communes, intercommunalités, juste à la fin, on a parlé des départements, moi je suis personnellement très sensible à la situation des départements qui sont dans une situation difficile et le 3ème chantier confié à la mission Richard Burr c'est justement sur les allocations de solidarité individuelle de solidarité nous savons comment les départements sont dans des situations difficiles, c'est pour ça qu'il y a eu dans le PLFR une enveloppe de 100 millions d'euros, ça n'est jamais suffisant, bien évidemment, mais ça va permettre à à peu près 25 départements les plus difficilement toucher d'avoir quand même bouffée d'oxygène, si je puis dire, pour pour faire face aux difficultés financières dans lesquelles ils sont nous sommes très attentifs il y assure à cette situation je crois qu'il faudra pour les départements, là aussi trouvé dans le la réforme des films de la fiscalité locale, de nouvelles ressources, je vous remercie. merci, madame la ministre, donc nous allons maintenant procéder à l'examen des amendements portant sur les crédits de la mission, relations avec les collectivités territoriales figurant donc à l'État B. alors le premier amendement est l'amendement 80 rectifié présenté par Madame Sylvie Robert. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, vous avez entendu le président de la République, faire de l'ouverture, et notamment de l'extension de Arthur des bibliothèques, une de ses priorités en matière culturelle, on sait qu'aujourd'hui les des biotechs sont effectivement un maillage très important sur notre territoire en termes d'équipements, c'est aujourd'hui le 1er équipement culturel publics de notre pays, la ministre de la culture pour traduire l'ambition du président a même nommé Erik Orsenna, vous savez, qui fait un tour de France et qui est un ambassadeur justement auprès des collectivités pour que, hé bien, les maires et les présidents des conseils départementaux, notamment pour les BTP puisse être encouragé à augmenter les horaires d'ouverture de leur bibliothèque c'est une très bonne chose par ailleurs. Se pose du coup la question du financement depuis plusieurs années, nous le savons, en tant qu'élus locaux, nous bénéficions pour aider à l'investissement des bibliothèques, nous, nous, nous bénéficions d'une aide de l'État, qui s'appelle la DG dès le concours particulier qui est au ministère de l'Intérieur depuis peu de temps cette DGB peut être fractionné pour pouvoir, justement, avoir de l'argent au fonctionnement parce qu'on sait que les horaires d'ouverture, c'est forcément de la masse salariale supplémentaire, donc forcément c'est du fonctionnement en matière de bibliothèques pour élargir les horaires d'ouverture des bibliothèques, je vous propose mes chers collègues, que cette DG des qui n'a jamais augmenté depuis plusieurs années et qui émane d'ailleurs a sensiblement diminué ces derniers temps, puisse être augmentée de 5 millions d'euros à la fois pour traduire l'ambition du président de la République, mais également pour pour cette dotation supplémentaire puisse aider les mères et les encourager à augmenter les horaires d'ouverture en ne pénalisant pas l'investissement qui est quand même encore la la la Terre vention de l'État, la plus significative, donc pour toutes ces raisons, mais, chers collègues, je vous demande de passer de 80 millions d'euros à 85 millions d'euros, ce qu'on appelle le concours particuliers la DGB merci.

oui madame la sénatrice donc vous nous proposez d'augmenter ses crédits, les crédits en faveur des bibliothèques municipales et départementales de 5 millions l'article 168 de la loi de finances pour 2016 a permis le financement par la DG comme vous l'avez indiqué de l'extension de l'évolution des horaires d'ouverture des bibliothèques municipales et départementales de près, via un concours particuliers qui effectivement est de 80,4 millions en en 2018: il est d'ailleurs stable, la majoration du crédit prévu par cette amendement nous semble prématuré alors que la réflexion lancée par le ministre de la culture sur ce sujet n'a encore pas abouti et le coût d'une éventuelle extension des horaires d'ouverture des bibliothèques n'est pas pour l'instant, chiffré par ailleurs la l'amendement cette augmentation par une ni Benusilho des crédits consacrés aux aides exceptionnelles aux collectivités territoriales, ce qui me gêne un peu, enfin cette possibilité ne revêt aucune caractère aucun caractère obligatoire et relève de la seule décision des collectivités territoriales concernées alors pour l'instant, nous avons un avis défavorable sur cet amendement. Merci de du gouvernement, Madame la Ministre. Madame la sénatrice Sylvie Robert, je sais que vous avez été l'auteur d'un rapport sur l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques dont Monsieur Éric Hersen, chargé d'une mission sur le sujet, nous avons eu connaissance d'un arbitrage du président de la République, augmentant la DG des bibliothèques de 8 millions d'euros pour accompagner les communes dans la mise en oeuvre

je vais vous demander de retirer votre amendement car cette augmentation ne-ce pas ne peut pas être financée comme vient de le dire, le rapporteur de la commission des lois sur la mission RCT, vous avez entendu suffisamment ici les intervenants et donc cette augmentation sera financé par le budget général et donc, je vous remercie, si vous acceptez de retirer votre amendement. Madame Robert. Eh bien écoutez, madame la ministre, je n'en attendait pas tant puisque nous devenons d'avoir quand même un arbitrage en seulement favorable mais une nouvelle qui va satisfaire, je pense, les maires et les présidents de conseils départementaux en matière de dos d'horaires d'ouverture, et notamment de leur bibliothèque bien évidemment je vais retirer mon amendement et bien évidemment, alors même que je l'avais gagé mais c'était au bénéfice des collectivités territoriales, puisque nous devons le faire je me réjouis de cette nouvelle par le président de la République et je pense que donc ce chantier est bien entamée, merci beaucoup. Merci, merci, donc l'amendement le 99 rectifier madame a-t-elle. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous avons beaucoup débattu avant l'été sur la réserve parlementaire dans le cadre de la loi pour la confiance dans la vie politique avant qui, si elle ne choix et surtout à l'Assemblée nationale au nom de la transparence et du clientélisme à cette occasion, nous avions ici au Sénat, évoqué l'incongruité du maintien de la réserve ministérielle qui procède d'une distribution pour le moins extrêmement discret mais sa suppression avait alors été adopté, toutefois, cette disposition a été déclarée inconstitutionnelle au nom de la séparation des pouvoirs, alors aujourd'hui nous souhaitons offrir au gouvernement l'occasion de pratiquer la vertu qu'ils nous recommandent et de concrétiser son attachement à nos collectivités en proposant cet amendement qui permettrait d'affecter des crédits de la réserve ministérielle du ministère de l'Intérieur en crédits pour nos collectivités, je vous remercie.

le Conseil constitutionnel, comme vous l'avait également rappelé, a estimé que cette mesure était contraire néanmoins si juridiquement la réserve ministérielle existe toujours, elle n'a pu être abondé dans le présent projet de loi de finances n'est pas abondé donc il y a sans doute un reliquat des décisions passées, mais il n'y a pas d'amendement nouveau, donc il n'y a pas aujourd'hui de création et donc cet amendement étant satisfait je demanderai donc aux auteurs de le retirer défendu seraient défavorables. vis à vis du gouvernement, Madame la Ministre. Madame la sénatrice Françoise-t-elle, il y a eu un avis effectivement du conseil constitutionnel et je vous rappelle que l'avis du Conseil constitutionnel, c'était que l'interdiction de la réserve ministérielle qui a été jugé inconstitutionnelle, c'est l'interdiction. ça veut dire quoi que. Ce n'était pas l'existence de la réserve ministérielle qui était inconstitutionnelle. Je croyais qu'il fallait le préciser néanmoins les crédits de la réserve ministérielle sont déjà supprimé, seuls sont prévues au PLF les crédits de paiement nécessaires pour les subventions déjà accordées dans les années passées, pour les opérations dont l'exécution se poursuit en 2018, il en est d'ailleurs exactement de même pour la réserve parlementaire aucune autorisé en notion d'engagement n'est inscrit, et donc il n'est plus possible d'attribuer de nouvelles subventions au titre de la réserve ministérielle comme autre petit de la réserve parlementaire et c'est une décision donc du du gouvernement. j'vais dire est-ce que vous maintenez l'amendement ou le retirer. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, et mes chers collègues, le rapporteur, je vous remercie de vos explications, je suis heureuse d'avoir déposé mon amendement qui a le mérite de clarifier les choses, que nous n'avions pas forcément eu la suite des épisodes de cette longue série de la mise en place d'un esprit vertueuse madame la Mini, je vous félicite de l'esprit vertueux qui est devenue très contaminant, et au vu des explications, je suis heureuse de vous faire plaisir en retirant mon amendement, puisque, semble-t-il, nous devons tous être heureux de la situation, je vous remercie. Merci, merci, donc les 2 amendements ayant été retirée, nous avons, nous allons procéder au vote des crédits de la mission, relations avec les collectivités territoriales figurant donc à l'État B. sachant que les parlementaires ne peuvent plus s'exprimer, ayant épuisé leur temps de parole en introduction, donc il n'y a pas d'explication de vote mais la Commission peut effectivement intervenir, de même que le gouvernement Monsieur Charles gagner. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, avant de voter sur les crédits de la mission, je voudrais rappeler les raisons qui ont conduit à la commission des finances à vous proposer des adopté cette session budgétaire, a été l'occasion d'examiner plusieurs dispositions qui suscitent des inquiétudes concernant les finances des collectivités locales, je pense à la trajectoire des dépenses à la contractualisation au mécanisme de correction à la nouvelle règle d'or à la suppression progressive de la taxe d'habitation à la minoration de la desserte épées et des fonds départementaux de taxe professionnelle à la suppression d'une part des crédits de la dotation d'action pas complémentaire destinée aux collectivités locales, etc, sur l'ensemble de ces points, le Sénat a corrigé le texte du gouvernement la trajectoire des dépenses a été modifiée dans un sens plus réaliste et plus favorable aux collectivités le mécanisme de contractualisation et de correction a été complété par un un bonus la nouvelle règle d'or a été supprimé, la réforme de la taxe d'habitation a été reportée en attendant qu'aboutissent, une réflexion plus large sur l'avenir de la fiscalité locale

c'est pourquoi la commission des finances, vous invite à adopter les crédits de la mission qui comprennent essentiellement des compensations de transferts de compétences et des dotations d'investissement.

y a pas de Madame la ministre, tout à fait, donc je vais mettre aux voix, les crédits de de la mission. Qui est pour.

Qui est contre. Merci qui s'abstient. Donc les les crédits sont adoptés, ce n'est pas l'abstention qui l'emporte, crédits adoptés donc je vais suspend la séance, elle sera reprise à 14 heures pour l'examen des articles rattaché à cette mission et les crédits du compte spécial avant ce collectivités territoriales, la séance est suspendue.